Parmi ces victimes, 11 % des femmes et 7 % des hommes ont déclaré des attouchements du sexe, 95 % des femmes des attouchements des seins ou des fesses, des baisers imposés par la force ou du pelotage, et 93 % des hommes du pelotage. Entre 20 et 34 ans, les agressions sexuelles touchent une femme sur vingt, soit cinq fois plus qu'entre 50 et 69 ans. La famille et l'entourage proche constituent un espace privilégié de victimation. Ainsi, 5 % des femmes y ont subi au moins une agression depuis leur enfance et 1,6 % au moins un viol ou une tentative de viol.

Les femmes subissent viols et agressions sexuelles dans de bien plus grandes proportions que les hommes. Pour elles, les violences dans le cadre des relations conjugales s'ajoutent aux violences subies au sein de la famille dès l'enfance et l'adolescence, ainsi qu'aux agressions tout au long de la vie, au travail ou dans l'espace public.

Certes, depuis vingt-cinq ans, un travail considérable a été accompli par les associations féministes et de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Depuis 2011, des plans gouvernementaux triennaux de lutte contre les violences faites aux femmes ont été lancés, ainsi que, en 2013, une mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains, la MIPROF. Sur le terrain, pourtant, ces initiatives n'ont pas bouleversé la donne. La loi du silence, le déni, l'impunité des agresseurs, l'abandon des victimes

Si vous voulez savoir pourquoi je n'ai rien dit, il vous suffira de chercher ce qui m'a forcé à me taire. [ ...] Si je vous dis ce qui m'est arrivé, vous n'allez pas me croire, vous allez rire, vous allez prendre le parti de mon agresseur, vous allez me poser des questions obscènes ou, pire même, vous aurez pitié de moi. [

pour ne pas être méprisé et pour se protéger lui-même en préservant son image. » Notre société continue de méconnaître la réalité des violences sexuelles, leur fréquence, la gravité de leur impact et de les reléguer dans la catégorie des faits divers. Cette méconnaissance participe à la non-reconnaissance des victimes et à leur abandon sans protection ni soin. Ce système, organisant le déni et la mise en cause des victimes elles-mêmes, qui auraient provoqué le viol ou l'agression sexuelle par leur comportement, a un nom : la « culture du viol ». Une société dans laquelle une part importante de la population estime que forcer sa conjointe ou sa partenaire à avoir un rapport sexuel alors qu'elle le refuse et ne se laisse pas faire n'est pas un viol, que forcer une personne à faire une fellation alors qu'elle le refuse et ne se laisse pas faire n'est pas un viol, ou encore qu'à l'origine d'un viol il y a souvent un « malentendu », est une société dans laquelle les victimes de violences sexuelles révélant ce qu'elles ont subi courent le risque d'être mises en cause et maltraitées. Comment attendre d'elles qu'elles parlent ? Or céder, faut-il le rappeler, n'est pas consentir. Maintes contraintes physiques, morales ou économiques peuvent permettre à une personne d'imposer des actes ou des comportements sexuels à une autre qui ne les veut pas, mais les subira sans mot dire ni s'opposer. La vision stéréotypée des violences sexuelles, parasitée par la « culture du viol », n'est pas seulement le fait des hommes

d'encourager les victimes à parler, pour les aider à sortir plus tôt de leur traumatisme. Pour 72 % des Français et des Françaises, les victimes de viol

Plus de deux Français sur trois jugent impossible de se remettre d'un viol.

Elle est de lancer des campagnes visant à améliorer, au sein de la population, la connaissance de la loi, des droits et des chiffres des violences sexuelles, ainsi qu'à déconstruire les représentations fausses qui portent préjudice aux victimes.

et le couple, mais aussi les institutions, les lieux publics, dont les transports en commun, et l'internet. Il est tout aussi impératif de mieux former les professionnels susceptibles d'être en contact avec les victimes : médecins, policiers, juges,

Elle exige que l'on donne aux médias les outils nécessaires pour qu'ils cessent de participer à la diffusion de représentations sexistes, de stéréotypes et d'idées fausses concernant les violences sexuelles. On sait qu'une proportion élevée d'enfants et de jeunes adolescents subissent des violences sexuelles. Ils devraient être prévenus des dangers qu'ils courent, apprendre comment et par qui ils peuvent en être protégés. Il ne faut jamais se lasser de répéter que leur protection passe avant celle de l'agresseur, avant celle, aussi, des intérêts et de la réputation de la famille, des institutions ou de la société, quand les mis en cause les mis en cause sont des personnalités publiques connues. Il paraît indispensable, à cet égard, d'inclure un volet relatif à la prévention des violences sexuelles dans la formation initiale des directeurs d'école, en l'inscrivant dans un projet éducatif plus global de promotion de la santé, élaboré avec les différents acteurs concernés au sein de l'école, en accordant une plus grande place à la parole de l'enfant et en établissant de bonnes relations avec les familles. esprit, l'accompagnement des enseignants dans la mise en oeuvre de la prévention passe par une réflexion sur le choix des pratiques pédagogiques. Malgré les efforts déjà déployés, le chemin est encore long. Nous sommes loin d'avoir rompu avec la « culture du viol ». Il ne s'agit pas seulement d'un travail institutionnel, mais aussi d'une démarche à conduire avec avec chaque victime, pour libérer sa parole de souffrance avant qu'elle ne se laisse envahir par elle, parfois pour des décennies. Il revient à chacun, là où il vit et là où il oeuvre, et à la société tout entière, au nom de la solidarité, de s'investir dans ce combat, pour rendre définitivement inacceptables les violences sexuelles et aider celles et ceux qui les subissent à sortir de leur silence, pour pouvoir se reconstruire. C'est aussi à sa capacité de mener pareil combat qu'une société démocratique comme la nôtre est jugée. La parole

de janvier, l'académie des Césars annonçait en grande pompe sur Twitter que le réalisateur franco-polonais Roman Polanski, 83 ans, présiderait la quarante-deuxième cérémonie des Césars, le 24 février prochain. L'industrie du spectacle, qui n'aime rien tant que les anniversaires, choisissait Roman Polanski quarante ans exactement après qu'il eut été accusé de viol sur une jeune fille de 13 ans, ce qui l'avait poussé à fuir les États-Unis peu après s'être déclaré coupable de « rapports sexuels illégaux Depuis, sous la pression des associations féministes, le réalisateur, dont personne ici ne nie le talent, a décidé de renoncer.

de culture dans notre pays. » Si le monde de la culture absout des agresseurs sans nuance ni scrupule, au prétexte qu'ils débordent de talent, comment la société peut-elle espérer que les victimes, confrontées à de telles amnisties, libèrent leur parole ? Car c'est un fait malheureusement avéré : très souvent, les victimes ne portent pas plainte parce qu'elles éprouvent un sentiment de honte ou de culpabilité, et elles s'enferment malgré elles dans cet état, parfois aussi pour épargner leurs proches. Elles craignent d'être tenues pour responsables de ce qui leur est arrivé, qu'on les soupçonne d'avoir été consentantes. C'est la funeste « culture du viol en raison de laquelle, pendant longtemps, les questions de la pédophilie, du viol ou des agressions sexuelles ont été peu abordées, pour ne pas dire taboues.

portant sur les représentations du viol et des violences sexuelles chez les Français donne des résultats effarants : 40 % des personnes interrogées estiment que la responsabilité du violeur est atténuée si la victime a eu une attitude provocante en public

Ces chiffres donnent la mesure du travail de pédagogie et d'accompagnement restant à accomplir. Selon le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, en moyenne

Mais, parmi ces personnes, 12 % seulement déposent plainte et seule une plainte sur dix aboutira à une condamnation. Ces données alarmantes font dire à la présidente du Collectif féministe contre le viol que, « dans le viol, la parole est le premier tabou ». À ce titre, l'accueil des victimes est le premier enjeu. Si, dès ses premiers mots, une victime a le sentiment qu'elle n'est pas crue, que l'accueil manque de confidentialité et n'est pas bienveillant, elle renonce à porter plainte. Pour remédier à cette situation, les policiers et gendarmes qui le souhaitent peuvent, depuis le début des années 2000, bénéficier d'une formation relative à l'accueil et à l'audition des femmes victimes de violences sexuelles.

ces professionnels est en effet capitale pour les victimes, et c'est aussi grâce à eux que de nombreuses femmes parviennent à aller au bout du processus et à se reconstruire. La présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, Danielle Bousquet, rappelle d'ailleurs que, en la matière, si des progrès indiscutables ont été faits, « il faut [ ...] aller plus loin, en s'inspirant de l'expérience de la cellule d'accueil d'urgence des victimes d'agressions du CHU de Bordeaux : les victimes peuvent y accéder en direct, c'est-à-dire sans dépôt de plainte préalable.

Ce dispositif est complété par les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, dont la mission est de venir en aide aux victimes d'agressions sexuelles, particulièrement en les accompagnant durant tout le processus judiciaire si elles décident de déposer une plainte. On le voit, la France gagnerait à s'inspirer de l'exemple du Québec, lequel a institutionnalisé l'ensemble du processus de prise en charge et d'accompagnement des démarches judiciaires, afin de sécuriser les victimes

les personnels de terrain savent souvent identifier les situations, comprendre les rapports de force et deviner les problèmes. Ce sont eux, et seulement eux, qui seront à même de définir si la personne a été ou

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

Après ces révélations, l'animatrice a dû faire face à des accusations de diffamation. Une partie de l'opinion l'a même accusée d'être responsable de la mort de l'auteur présumé Cet enchaînement de faits révèle, en raison de la notoriété des protagonistes, ce que vivent dans l'ombre des milliers, voire des millions, de victimes de violences sexuelles : l'horreur du drame et ses conséquences tout au long de la vie, la difficulté, voire l'impossibilité, d'en parler, d'être crue, le déchaînement de violences, de ruptures auquel de nombreuses victimes ont à faire face lorsque leur parole se libère. preuve, s'il en était besoin, que notre société n'entend pas ces victimes, pour plusieurs raisons. Le huis clos dans lequel se déroulent ces abus et ces crimes muselle la parole des victimes. La violence physique et psychologique, la peur rendent le crime presque parfait, car l'enjeu pour l'auteur des faits, en plus d'abuser sexuellement sa victime, est d'empêcher la parole

Je tiens à saluer à mon tour l'initiative de mes collègues du groupe écologiste. L'enjeu est fort. La parole est le point de départ de la reconstruction des victimes et le point d'arrêt des criminels. Encore faut-il que la société accepte de regarder, d'écouter cette réalité et de mettre en oeuvre les moyens d'accompagner cette parole, de la rendre audible. Au-delà de la révélation, il s'agit de proposer des lieux de réparation. Commençons par regarder les choses en face : les violences sexuelles, qu'elles s'exercent sur des enfants ou sur des adultes, sont un phénomène d'ampleur dans notre pays.

d'une plainte. Le Conseil de l'Europe estime qu'un enfant sur cinq est confronté à la violence sexuelle sous toutes ses formes : viols, abus sexuels, pornographie, sollicitation des enfants par le biais d'internet, prostitution et corruption. Selon le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'âge de 20 ans, une Française sur dix déclare avoir été agressée sexuellement au cours de sa vie, dans le cercle familial pour la très grande majorité d'entre elles. Ces chiffres sont effrayants. Ce matin, nous parlons d'un type de violences bien spécifique, les violences sexuelles, mais je souhaite insister sur le fait que ces violences s'inscrivent dans un contexte social très permissif. Les auteurs se sentent tout-puissants, ce qui décourage les victimes de parler. On peut évoquer un des violences au niveau individuel et au niveau collectif. Au niveau individuel, toutes les violences subies dans l'enfance meurtrissent, abîment profondément. Les violences sexuelles sont encore plus La victime risque, plus que toute autre personne, d'être surexposée à d'autres violences à l'école, et plus tard au sein du couple ou au travail. Elle risque aussi de développer des comportements à risque contre elle-même ou contre les autres. Si la victime n'est pas prise en charge, elle peut souffrir de ce de violences tout au long de sa vie. Nous retrouvons ce au niveau sociétal, car même si les garçons et les hommes sont aussi victimes de violences, sexuelles notamment, celles-ci s'inscrivent toujours dans un contexte de domination sexué. Les auteurs sont très majoritairement des hommes, et les victimes sont majoritairement des femmes et des enfants. Toutes les formes de violences se conjuguent et se renforcent

On peut aussi évoquer un chez les auteurs de violences. Violaine Guérin, endocrinologue et gynécologue médicale, présidente de l'association Stop aux violences sexuelles, indique, en s'appuyant sur les travaux de la psychanalyste Alice Miller, que « la violence est racine de est racine de la violence ». Elle avance même que 80 % des agresseurs auraient eux-mêmes subi des abus dans leur enfance. Il y a donc urgence à traiter ce fait social, de santé publique que sont les violences sexuelles, en agissant au niveau individuel et au niveau collectif. La politique conduite ces dernières années en matière d'égalité entre les femmes et les hommes a permis de mettre en évidence, de mesurer les inégalités et de rechercher des moyens d'atteindre l'égalité réelle. des avancées, il reste beaucoup à faire. Nous devons centrer nos efforts sur les droits des enfants et opter pour une éducation bienveillante. Il faut informer davantage les mineurs sur leurs droits.

Son article 222, que les deux chambres avaient enfin fini par adopter, disposait que l'autorité parentale s'exerce à l'exclusion de « tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles Cette censure, pour une question de forme, permet à certains parents de continuer à user d'un archaïque « droit de correction » sur leurs enfants. C'est bien regrettable Au niveau individuel, il s'agit de créer un climat de confiance propice à la libération de la parole de la victime, de croire celle-ci et de l'accompagner. Comme nous l'apprennent de nombreux témoignages, il est tout d'abord difficile de faire émerger ces événements à la conscience : la victime les enfouit pour survivre. On parle d'amnésie traumatique. Ce travail personnel peut prendre de nombreuses années, voire ne jamais se faire. La victime doit affronter la honte et l'emprise, mécanismes spécifiques aux agressions sexuelles. la question est « en parler ou non ». En effet, pour les personnes victimes de violences sexuelles, le fait même d'en parler constitue une expérience redoutable. En parlant, en déposant plainte, elles vont revivre les épisodes douloureux. Elles prennent le risque de se retrouver face à leur agresseur, d'être exclues de leur famille, accusées de mensonge, menacées de mort. Pour tenir, il faut impérativement être accompagné. Cet accompagnement pourrait être assuré au sein de centres de crise et de soin spécifiques et pluridisciplinaires pour les enfants et les adultes victimes de violences sexuelles, comme le propose la psychiatre Muriel Salmona des lieux de soins, mais aussi des lieux ressources pour les intervenants professionnels et bénévoles. Dans les cas où les faits ne sont pas prescrits, c'est alors « parole contre parole ». La victime s'expose à une nouvelle charge de violence de la part de l'agresseur. En l'absence de preuves, comme c'est très souvent le cas pour ces faits, le dossier est classé sans suite. La victime n'a pas obtenu la reconnaissance attendue. Parfois, lorsque les faits sont prescrits, le dépôt de plainte permet la découverte de nouvelles victimes, pour lesquelles les faits peuvent être

En témoignant, elle risque d'être poursuivie pour diffamation ; c'est inique ! Devant un fait social d'une telle ampleur, il faut prendre les moyens d'aider les victimes à se réparer. est essentiel de former les professionnels et les bénévoles à la réalité des violences sexuelles, à leur ampleur, à leurs mécanismes de destruction et à la reconstruction de la personne, que ce soit dans le champ médical, dans l'éducation ou dans le monde du travail. Par ailleurs, nous devons poursuivre les travaux engagés ici sur l'initiative de notre collègue Colette Giudicelli en instaurant une obligation de signalement pour le personnel médico-social qui repère des violences sexuelles chez un patient. Aujourd'hui, une vision conservatrice demeure au sein des ordres médicaux, qui, sous couvert de respect du secret professionnel, s'opposent à l'obligation de signaler. Si, à l'automne 2015, nous avions réussi à faire en sorte que le signalement ne puisse se retourner contre le soignant, nous devons aller plus loin, en assurant la confidentialité des informations transmises. En effet, dans certaines situations, le signalement profite à la défense du mis en cause, par exemple quand celui-ci est détenteur de l'autorité parentale et peut donc consulter les dossiers relatifs à la victime

Pour conclure, mes chers collègues, je me réjouis que ce débat ait lieu. Il nous honore. Ces dernières semaines, en effet, nous avons pu entendre dire que députés et sénateurs se désintéressaient de la question des violences sexuelles. Il n'en Il n'en est rien. Nous continuons le combat en faveur des victimes. Nous voulons une société plus juste, plus respectueuse de chaque être humain. Continuons à dénoncer toutes ces formes de violences. Je pense notamment à un phénomène récent, celui des « viols à distance », sur commande et par internet, qui se répandent dans les réseaux pédophiles. Continuons aussi à dénoncer toutes les inégalités et injustices desquelles se nourrissent toutes ces violences. Rien n'est inéluctable, et l'intervention de la loi en la matière est déterminante pour signifier quelle société nous voulons construire. La mobilisation de l'opinion publique, les prises de position de personnalités du monde du spectacle, aux côtés de la comédienne Andréa Andréa Bescond, en faveur de l'imprescriptibilité, nous interpellent et nous servent d'aiguillon. Soyons attentifs à la souffrance des victimes

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui, sur l'initiative d'Esther Benbassa, pour aborder le délicat sujet des violences sexuelles et de la nécessité d'aider les victimes à en parler. Je voudrais remercier le groupe écologiste de nous permettre d'avoir ce débat difficile mais ô combien utile. En effet, même s'il est difficile d'avoir des chiffres fiables et représentatifs, une femme sur cinq et un homme sur quatorze interrogés dans le cadre de consultations médicales déclarent avoir déjà subi des violences sexuelles. En se fondant sur les seuls dépôts de plainte, on peut estimer que près de 260 000 personnes seraient chaque année victimes de viols ou tentatives, dont plus de 125 000 filles et 32 000 garçons de moins de 18 ans, selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes.

Une sur deux avait moins de 11 ans, une sur cinq moins de 6 ans. Dans 96 % des cas, l'agresseur est un homme. Un enfant victime sur deux est agressé par un membre de sa famille. Dans un cas sur quatre, l'agresseur est lui-même mineur. Je rappelle que, à l'âge adulte, un viol sur deux serait un viol conjugal. Seulement 18 % des viols de personnes majeures seraient le fait d'un inconnu.

Ce rapport dresse une longue liste des pathologies somatiques associées aux violences sexuelles. En touchant à l'âme des victimes, les agresseurs font aussi des ravages dans leur corps. Plusieurs études scientifiques ont montré qu'avoir subi de tels faits serait un facteur de risque, parfois plusieurs décennies après, de développer des maladies cardiovasculaires, pulmonaires, endocrines, auto-immunes, neurologiques, des problèmes de sommeil et de douleurs chroniques, voire des atteintes épigénétiques pouvant être transmises à la descendance des victimes. Les conséquences sont encore plus graves quand l'agression était incestueuse : plus la victime est jeune au moment des faits, plus l'agresseur est proche d'elle, plus il a d'autorité sur elle, et plus l'impact sur sa qualité de vie et le risque qu'elle tente de se suicider sont importants, nous disent les professionnels. L'abus reste un secret absolu très longtemps, parfois toute une vie. En gardant le silence, la victime se fait, malgré elle, l'alliée de l'abuseur, puisque la seule chose que celui-ci redoute, c'est d'être dénoncé. Le fait de devenir ainsi, bien involontairement, son alliée, renforce le mépris que la victime a d'elle-même et son sentiment Pourtant, une personne sexuellement abusée n'est jamais coupable ni responsable. Mais parler est pour elle très difficile, peu de victimes portent plainte. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics d'aider à améliorer la prise en charge et l'accompagnement des victimes. Seules 4 % des victimes agressées dans l'enfance disent avoir été prises en charge par l'aide sociale à l'enfance, 70 % de ceux qui ont porté plainte pour des faits commis alors qu'ils étaient mineurs n'auraient jamais été protégés et que 70 % de l'ensemble des victimes se sont senties insuffisamment ou pas du tout reconnues comme telles. C'est pourquoi la prise en charge médicale doit être améliorée, afin qu'elle soit plus rapide et mieux adaptée à l'état de stress post-traumatique victimes. Ces enseignements figurent au programme des épreuves classantes nationales d'accès à l'internat, mais de nombreux étudiants interrogés semblent l'ignorer. En effet, alors que 30 % d'entre eux ont été confrontés aux violences sexuelles moins d'un sur cinq indique avoir déjà reçu un cours ou une formation sur ce sujet, à l'issue de la réforme menée en 2012-2013. À ce jour, ces troubles restent mal diagnostiqués par les médecins. Ils sont souvent mis sur le compte de troubles de la personnalité, d'une dépression, voire d'une psychose. santé, l'OMS, avoir subi des violences sexuelles est le facteur de risque principal d'en subir à nouveau ... C'est pourquoi il faut libérer la parole. Un important travail d'information est d'ores et déjà mené auprès des personnes sexuellement violentées, notamment par les associations, qui sont très présentes et dont je tiens à souligner l'extraordinaire travail. Idéalement, il faudrait réussir à créer, dans chaque ville moyenne, une consultation spécialisée en psycho-traumatismes associée à un réseau de professionnels formés et informés.

Je suis convaincue que, pour combattre ce fléau, il ne faut pas opposer ceux qui sont chargés du sujet et ceux qui ne le seraient pas. Il y a urgence à sensibiliser tous les professionnels qui sont en contact avec les enfants,

Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons endiguer ce fléau et aider les victimes à parler ! La parole

Le sujet est grave et complexe : il touche à l'humain, à son intimité, à ses souffrances les plus terribles. Ce débat Ce débat doit être consensuel. Il nous faut agir ensemble contre ce fléau qui frappe aussi bien des femmes et des hommes que des enfants. Nous devons faire front dans l'intérêt de nos concitoyens. Dans notre pays, une femme sur cinq et un homme sur quatorze déclarent avoir subi des violences sexuelles. Dans 94 % des cas, les agresseurs sont des proches, parfois même des membres de la famille, hélas ! Très peu de victimes portent plainte, par honte, par crainte, par pudeur, par peur de détruire la cellule familiale. À la lumière de ces chiffres alarmants, on comprend très bien quel est

de violences sexuelles en matière de prescription, nous devons également nous pencher sur les dispositifs nécessaires à la libération de la parole. L'impunité et le silence ne doivent jamais être la règle. Notre pays doit nécessairement renforcer tous les dispositifs de prévention au bénéfice des personnes les plus exposées, expliquer où se situent les limites de l'acceptable, diffuser un message de tolérance zéro à l'égard des actes odieux et encourager la parole. la parole. Sortir du silence permettra aux victimes de mieux se reconstruire. L'accompagnement des victimes et de leurs familles doit être renforcé pour éviter tout enfermement et, surtout, toute culpabilisation. La justice doit avoir les moyens de remplir pleinement son rôle et de sanctionner, au nom de la société, ces actes odieux. Il faut commencer par faire de la pédagogie en milieu scolaire, et ce dès le cours préparatoire. C'est un bon moyen de prévenir l'installation d'un silence souvent dévastateur. Les violences sexuelles sont traumatisantes. Certaines et certains n'en parlent que difficilement, seulement avec l'aide d'un thérapeute. D'autres n'y arrivent jamais.

La force physique, quant à elle, n'est pas nécessairement employée dans les violences sexuelles : c'est la raison pour laquelle il n'en résulte pas toujours des traumatismes physiques. Les atteintes à la santé génésique, à la santé mentale et au bien-être social comptent parmi les conséquences les plus courantes de la violence sexuelle. Une étude française portant sur des adolescentes conclut également à l'existence d'un lien entre le fait d'avoir été violée et l'apparition de troubles du sommeil, de symptômes de dépression, de plaintes somatiques, la consommation importante de tabac et certains troubles du comportement courant, comme le fait d'avoir une attitude agressive. Ces manifestations sont propres à chaque victime et varient avec le temps. C'est pourquoi la victime doit être aidée et accompagnée de façon très personnalisée. Il me paraît essentiel que nous débattions de l'importance des approches individuelles. Les soins et le soutien psychologique, par l'intermédiaire de conseils, d'une thérapie et de groupes de soutien, se révèlent utiles après des agressions sexuelles, surtout lorsque le processus de rétablissement est compliqué. Certains faits montrent qu'un programme de courte durée, alliant thérapies cognitive et comportementale, suivi peu après l'agression peut contribuer à une atténuation plus rapide du traumatisme psychologique subi. les victimes de violences sexuelles se sentent souvent responsables de ce qui leur arrive, et il est démontré qu'il est important, pour leur rétablissement, de traiter ce sujet en psychothérapie. Pour faire face à ce fléau dramatique, des actions concrètes doivent être mises en place. Nous devons en être les garants.

Dans d'autres pays, la télévision est utilisée efficacement pour alerter le grand public sur les violences sexuelles. À mes yeux, il est nécessaire d'accorder davantage d'attention à la prévention primaire de la violence sexuelle. Celle-ci est d'ailleurs beaucoup trop souvent négligée au profit des services aux victimes.

Il faut également améliorer la formation des policiers et des gendarmes, qui sont souvent les premiers interlocuteurs de la victime souhaitant dénoncer son agresseur. Si l'on n'a pas reçu une formation adaptée, il est difficile d'adopter le bon comportement pour ne pas brusquer ou inquiéter une victime déjà très fragilisée. Nos policiers et nos gendarmes se dévouent pour protéger nos concitoyens. Leur apporter ce type de formation va directement dans le sens de l'amélioration du service rendu à la population. La violence sexuelle est un problème de santé publique courant et grave, qui affecte des milliers de personnes chaque année en France. Elle est dictée par de nombreux facteurs qui agissent dans différents contextes économiques, sociaux et culturels. L'inégalité des sexes est au coeur de la violence sexuelle dirigée contre les femmes,

La séance est reprise. La parole est à Mme Laurence Cohen.

pour améliorer la prise en charge des victimes, pour mettre fin à ces violences. Nous devons donc étudier les obstacles sociaux et juridiques qui font qu'aujourd'hui, dans notre société, les victimes, adultes comme enfants, ont tant de mal à dénoncer leurs harceleurs et leurs agresseurs.

osent parler. Permettez-moi de faire un « focus » sur le viol, forme la plus extrême de ces violences, en reprenant les chiffres des ministères de l'intérieur et de la justice. 84 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de viol ou de tentative de viol. Moins de 10 % de ces femmes déposent plainte, et seule une plainte sur dix aboutit à une condamnation. 51 % des femmes victimes de viol ou de tentative de viol ne font aucune démarche, ni auprès des forces de police ou de la gendarmerie, ni auprès de médecins, psychiatres et psychologues, ni auprès des services sociaux, associations ou numéros d'appel. Ce sont là des chiffres, hélas ! relativement constants, qui ne diminuent pas au fil des années, malgré les politiques publiques déployées jusqu'à présent, notamment par vous, madame la ministre. Ce débat est donc bienvenu pour nous permettre de réfléchir ensemble aux mesures urgentes qu'il faut prendre, par le législateur comme par l'État. On ne peut analyser ces violences qui gangrènent notre société sans insister sur le caractère « genré » de ce fléau : la très grande majorité des victimes sont des femmes. Malgré les luttes menées par les féministes et les progressistes, le patriarcat est un système de domination qui continue d'imposer sa loi. Je tiens à dénoncer un premier obstacle qui empêche les femmes victimes de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle de parler, ou d'ailleurs de toute forme de violence : la honte, la culpabilité de ne pas avoir réagi et de devoir affronter incompréhension et jugement réprobateur.

Je pense bien sûr ici au cas de Jacqueline Sauvage, dans lequel cette dimension n'a été que trop peu prise en compte. Les travaux de Muriel Salmona démontrent également que les violences sexuelles accroissent fortement les risques de détresse psychologique et d'apparition de symptômes liés à un état de stress post-traumatique.

Il faut inverser la culpabilité et mettre un terme à cette forme de tolérance sociale des agressions sexuelles. Pour reprendre le slogan de l'association Osez le féminisme !, « la honte doit changer de camp Le second obstacle est le traitement que la justice réserve aux violences faites aux femmes, et singulièrement aux violences sexuelles. Comment ne pas dénoncer la longueur des procédures judiciaires ? Comment ne pas s'indigner que la parole des femmes soit remise en cause et que les faits soient le plus souvent minimisés ?

à souligner que les harceleurs et agresseurs se retrouvent dans tous les milieux sociaux professionnels, en zone urbaine comme en zone rurale. Oui ! Bien sûr, il faut encore améliorer et amplifier le travail mené auprès des agresseurs, dans un souci de prévention.

et d'éviter les délais trop longs. Le viol n'est pas un délit et ne doit donc pas être requalifié en agression sexuelle : c'est un crime, qui doit être jugé en cour d'assises. C'est très important ! Tout cela exige bien entendu que des moyens soient accordés à la justice,

de débarrasser la société des violences sexuelles et, plus largement, de toutes les violences faites aux femmes. C'est la condition à remplir pour conquérir l'égalité entre les femmes et les hommes. « Là où il y a une volonté, il y a un chemin », disait Lénine ! La parole

les hommes, les trois quarts des victimes étaient mineures au moment des faits et près des deux tiers avaient moins de 15 ans. En 2015, la moitié des victimes de violences sexuelles enregistrées par la police et la gendarmerie avaient moins de 15 ans. nous ne disposons d'aucune évaluation précise du nombre d'enfants victimes de violences sexuelles en France. En 2010, le Conseil de l'Europe avançait qu'un enfant sur cinq sur notre continent était victime de ces violences entendues au sens large : viols, tentatives de viol, agressions sexuelles, exposition à la pornographie, exploitation sexuelle et prostitution. Ces chiffres l'attestent, nous avons affaire à un phénomène de masse, certainement toujours sous-estimé pour ce qui concerne les plus jeunes. La loi du silence et le règne du déni en minorer encore l'ampleur, voire à le rendre invisible. L'absence de données fiables sur les violences sexuelles commises sur des hommes majeurs, qu'elles relèvent d'agressions homophobes ou qu'elles s'exercent en milieu carcéral, illustre bien

est donc un préalable à une prise en charge efficace. Là est l'enjeu majeur. Les sentiments de honte, de culpabilité, d'humiliation que ressentent toutes les victimes de violences sexuelles et qui sont entretenus par l'adhésion majoritaire de la société aux fausses représentations sur le viol

libérer la parole que, contrairement aux idées reçues, les viols et les agressions sexuelles se produisent majoritairement au sein du couple ou de la famille, au domicile de la victime, à son travail ou dans les institutions qu'elle fréquente. Cela a été rappelé, dans 90 % des cas, les violences sexuelles sont commises par une personne connue de la victime : le conjoint ou l'ex-conjoint pour près de 50 % des viols perpétrés sur des femmes adultes, un membre de la famille pour plus de la moitié des viols sur mineur. Pour les jeunes victimes, parler et être crues est un véritable défi. Outre la difficulté de reconnaître une agression sexuelle, de mettre des mots sur des actes insensés, d'identifier d'identifier un interlocuteur ou une interlocutrice à qui s'ouvrir, le poids du tabou de la violence sexuelle dans la sphère familiale pèse très lourdement sur la parole de ces enfants.

Ensuite c'est la crainte de faire mal à cette famille que l'on risque de faire voler en éclats. Et enfin c'est la honte de n'avoir finalement rien osé dire. Cette même honte qui nous fait nous sentir coupables, monstrueux et sales. Comment dire l'indicible ? Comment penser l'impensable ? Il est urgent de donner à toutes les victimes, et tout particulièrement aux plus jeunes d'entre elles, les moyens de signaler les violences qu'elles ont subies, et aux professionnels les outils pour recueillir leur parole de manière appropriée et respectueuse.

qui sont les premiers recours des victimes, s'est accru. Il s'agit de permettre aux professionnels de mieux repérer les violences. Travailleurs sociaux, personnels soignants, magistrats, fonctionnaires de police, gendarmes ou responsables associatifs ou responsables associatifs : tous, dans leurs fonctions respectives, sont des maillons essentiels d'une même chaîne. La cohérence et l'articulation de leurs interventions sont essentielles pour garantir aux victimes une prise en charge optimale. Il est donc impératif que toutes et tous disposent des mêmes repères et puissent s'approprier des outils communs. Quels que soient le professionnalisme, l'investissement et l'empathie dont chacun fait preuve, nul n'est à l'abri des préjugés, des interrogations ou des maladresses face à un phénomène qui doit être appréhendé dans toute sa complexité pour être traité de manière efficace. Poser les bonnes questions aux victimes, offrir un cadre d'écoute qui les aide à trouver les mots, leur rappeler qu'elles ne sont en rien responsables ou coupables de ce qu'elles ont subi : c'est le préalable indispensable pour libérer leur parole. Voilà pourquoi nous avons fait de la formation des professionnels

et un kit de constatation en urgence disponible dans les centres hospitaliers ; les magistrats peuvent suivre un stage de trois jours en formation continue à l'École nationale de la magistrature ; des modèles de certificats médicaux, élaborés en lien avec le conseil de l'Ordre des médecins, ont été mis en ligne sur le site internet de la MIPROF, ces certificats médicaux constituant des éléments de preuve obligatoires pour engager une action judiciaire ou permettre aux femmes de bénéficier d'une ordonnance de protection et, le cas échéant, d'un téléphone « grave danger ». Cette dynamique vertueuse est poursuivie et amplifiée au travers du cinquième plan

La loi du 14 mars 2016 a également contribué à accroître nos moyens en matière de protection de l'enfance et de détection des violences faites aux enfants.

de travailler ensemble dans le cadre des procédures d'enquête et constituent un lieu dédié, adapté et non anxiogène pour recueillir la parole de l'enfant et apporter les premiers soins nécessaires. Chantal Jouanno m'a interrogée sur l'instruction du 20 avril 2016,

en tant que personnalités qualifiées, par le biais d'une réquisition, en appui à un officier de police judiciaire. Sur les 1 774 militaires de la gendarmerie formés à l'audition de mineurs victimes, 3,7 % travaillent aujourd'hui au sein

comporte un volet spécifique pour renforcer l'accès aux droits et aux soins des jeunes filles et des femmes victimes de violences sexuelles. Fin 2016, le Gouvernement a engagé une large réflexion sur la prise en charge des traumatismes graves des adultes, des adolescents et des enfants victimes d'attentats. Les connaissances qui résulteront de ce travail de recherche-action de recherche-action seront mobilisables et transposables aux cas de violences sexuelles, en vue d'améliorer l'accompagnement des victimes, quel que soit leur âge. L'objectif est que chaque victime, où qu'elle réside, puisse bénéficier d'une prise en charge psychologique adaptée à la spécificité des psychotraumas, grâce à un maillage territorial renforcé des unités de soin.

L'enquête de l'IPSOS de mars 2016 sur les représentations du viol et des violences sexuelles révélait que 40 % des Français estiment que « la responsabilité du violeur est atténuée si la victime a eu une attitude provocante en public ». Il nous reste donc un travail important de déconstruction à mener ...

Enfin, la mobilisation « Sexisme, pas notre genre ! », qui vise à mettre en lumière la dimension systémique du sexisme, de la misogynie et de la domination